La séance est reprise. Les conclusions adoptées par la conférence des présidents réunie ce jour sont consultables sur le site du Sénat. Elles seront considérées comme adoptées en l'absence d'observations d'ici à la fin de la séance.-

Si le recours au contrat peut permettre d'ouvrir la fonction publique à un éventail de profils plus variés, il ne peut avoir pour conséquence de recruter des candidats moins qualifiés que ne le sont les fonctionnaires occupant un même poste.

qui est le syndicat majoritaire des enseignants du primaire, 775 recrutements manquent à l'appel à l'issue du concours, dont 361 à Créteil et 338 à Versailles.

ce qui est tout à fait satisfaisant. Toutefois, les solutions de mobilité ou de détachement de ces agents contractuels restent très limitées et sont souvent trop restrictives, que ce soit en termes de fonctions exercées- doivent être de même nature que les précédentes fonctions -, que de types d'employeurs, lesquels ne pouvant être que des collectivités publiques. Le présent amendement a pour objet d'élargir les possibilités de bénéficier d'une mise à disposition et de simplifier le dispositif, sans pour autant reconnaître aux contractuels des droits aussi importants

de la commission ? Cet amendement vise à élargir les conditions dans lesquelles les agents contractuels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics peuvent être mis à disposition d'une autre personne publique, voire d'une personne privée exerçant des missions de service public. Seraient concernés aussi bien les agents en CDI que ceux en CDD. Le projet de loi, tel qu'amendé par la commission, prévoit d'élargir les possibilités de recrutement par contrat dans la fonction publique territoriale, y compris en CDI. Toutefois, un agent contractuel n'est pas dans la même situation qu'un fonctionnaire. fonctionnaire. Il n'est lié contractuellement qu'à son employeur, alors qu'un fonctionnaire territorial est titulaire d'un grade qui lui donne vocation à exercer des fonctions dans toute collectivité. Un agent contractuel est recruté pour occuper un emploi spécifique, alors qu'un fonctionnaire a vocation, par le grade qu'il occupe, à occuper tous les emplois correspondants. Il nous est loisible de faire coexister, au sein des administrations, le système de l'emploi avec le système de la carrière, mais il ne faut pas confondre les deux, au risque de faire perdre toute attractivité aux concours de fonctionnaires. L'avis est donc défavorable.

Les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel les vacances de tout emploi dès qu'elles ont lieu. Seules certaines publications d'emploi particulières peuvent être réservées à des contractuels, telles que les emplois non permanents, notamment les remplacements d'agents absents

de la commission ? Le Gouvernement propose de supprimer l'article 6, introduit en commission sur l'initiative du groupe socialiste et républicain. Cet article prévoit qu'un avis de création ou de vacance d'emploi ne peut réserver cet emploi à un agent contractuel mais peut seulement indiquer qu'il est susceptible d'être pourvu par un contractuel.

L'indisponibilité d'un agent ne constitue pas une vacance d'emploi. Il n'y a donc pas lieu, dans ce cas, de publier un avis de vacance. La règle introduite en commission ne trouvera donc pas à s'appliquer. Nous n'avons pas non plus imposé, à l'article 6, la publication des créations d'emplois temporaires dans la fonction publique de l'État. L'avis est donc défavorable.

cet article est issu d'un amendement que nous avions déposé et qui a été adopté par la commission. Il prévoit qu'un emploi public ne puisse être strictement réservé à un contractuel, tout en étant évidemment

Mme Victoire Jasmin. Il s'agit par cet amendement d'encadrer les droits et obligations, notamment en matière de déontologie, des contractuels qui seront recrutés sur des emplois permanents au sein de la fonction publique.

De telles dispositions sont déjà prévues par les décrets propres aux agents contractuels des trois versants. Les modalités de recrutement et de travail des agents contractuels relèvent du domaine réglementaire, contrairement aux fonctionnaires titulaires,

Le Gouvernement propose de supprimer l'article 6, introduit en commission sur l'initiative du groupe socialiste, qui élève au niveau législatif les interdictions de recrutement d'agents contractuels liées aux condamnations antérieures. Les conditions de recrutement et d'emploi des agents contractuels des administrations des trois versants relèvent du domaine du règlement. J'observe cependant que le projet de loi comprend de nombreuses dispositions à ce sujet, ce qui a conduit la commission à faire preuve de mansuétude dans son appréciation de la recevabilité des amendements au titre de l'article 41 de la Constitution. Selon l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles relatives aux garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État et détermine les principes fondamentaux du droit du travail. si l'on fait une lecture stricte de ces dispositions, même les principes fondamentaux du droit applicable aux agents contractuels de droit public semblent échapper à la compétence du législateur. Il y a là une incongruité que nous pourrions être tentés de corriger à l'occasion d'une prochaine révision constitutionnelle. En réalité, il me semble que le développement du recours au contrat dans la fonction publique conduira nécessairement le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État à faire évoluer leur jurisprudence sur la ligne de démarcation entre la loi et le règlement en la matière. Il ne serait pas illogique que la compétence du législateur pour déterminer les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires soit étendue aux agents contractuels. De même, on pourrait plaider que la définition des conditions de recrutement d'agents contractuels relève des garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, au nombre desquelles certains auteurs rangent l'égal accès aux emplois publics. L'avis est donc défavorable.

Tout d'abord, la notion de condamnation pénale incompatible avec l'exercice de fonctions paraît trop vague pour les employeurs publics chargés de l'appliquer, de sorte que quelques jurisprudences sont venues clarifier les règles d'application des dispositions qu'il est prévu d'inscrire dans la loi. Je citerais notamment une décision n° 367724 du Conseil d'État en date du 4 février 2015, dans laquelle celui-ci confirme la décision d'un tribunal administratif ayant annulé la décision d'un directeur d'hôpital, au motif que ce dernier aurait commis une erreur d'appréciation en licenciant une employée agent d'entretien qui avait été condamnée pour complicité de transport, de détention, d'acquisition, d'offre ou de cession de stupéfiants, « en acceptant que soient conservés à son domicile des substances et des fonds liés au trafic » de son époux. Le directeur d'hôpital avait, dans la requête, invoqué un moyen tiré de risques pour la réputation de son établissement. Pour les agents titulaires, on observe également des cas d'annulation de radiations des cadres de la fonction publique territoriale d'agents après une condamnation pour des faits comme la conduite en état d'ivresse et le refus de se soumettre à un contrôle de police, pour des fonctions ne nécessitant pas la conduite d'un véhicule. Afin d'éviter que de telles erreurs d'appréciation ne se traduisent par de longues batailles contentieuses jusqu'au Conseil d'État, notre amendement vise à renforcer la proportionnalité de l'appréciation d'incompatibilité portée par les employeurs publics. Cela reviendrait à intégrer la jurisprudence du Conseil d'État au corpus législatif. Par ailleurs, une interprétation systématiquement large de cette incompatibilité par les employeurs publics aurait pour conséquence de nuire à la réinsertion sociale des personnes condamnées, étant rappelé que le service public représente un bassin d'emplois de 5,5 millions d'agents. Cela pourrait aussi considérablement nuire à la politique de réinsertion et, surtout, à la prévention de la récidive. Quel de cet amendement, Mme Delattre, propose de préciser que l'interdiction de recruter un agent contractuel frappé par une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions ne s'applique que si cette incompatibilité est manifeste.

Il est vrai que le Gouvernement a essayé de nous faire voter la suppression de l'article 6, ce que je n'ai pas fait puisque j'espérais que mon amendement serait adopté. Mais puisque Mme la rapporteur a l'air de dire que celui-ci est peut-être satisfait, je le retire.

est à M. Jérôme Durain. Cet amendement vise à créer, pour chacun des trois versants de la fonction publique, une règle de parité des rémunérations entre les fonctionnaires et les agents contractuels. Le Gouvernement justifie sa politique de suppression de postes de fonctionnaires par les contraintes budgétaires qui pèsent sur l'État et, au-delà, sur l'ensemble des employeurs publics. Mais à quelle logique répond le remplacement de fonctionnaires par des agents contractuels recrutés sur la base d'une rémunération plus élevée ? Au-delà de la vision court-termiste qu'illustre cette pente, et que le projet de loi tend à accentuer, ces divergences de rémunération entre fonctionnaires et agents contractuels au sein d'un même service pour un même type d'emploi est la source légitime d'incompréhensions et de tensions, nuisibles à la bonne marche du service public. Avec ce point, revenons à la question de l'attractivité de la fonction publique, que nous avons évoquée précédemment. Ce défaut d'attractivité, il faudra bien le monnayer s'agissant des non-fonctionnaires, c'est-à-dire des agents contractuels. Le même raisonnement prévaudra tout à l'heure quand nous aborderons la rupture conventionnelle. Un certain nombre de dispositions prévues dans ce texte et présentées comme des avancées auront des conséquences budgétaires pour les employeurs publics, pour les collectivités. Sur ce sujet, nous sommes donc assez offensifs en exigeant cette règle de parité.

Je n'y suis pas favorable. Ce serait contraire à notre tradition juridique, et cela priverait systématiquement les employeurs publics d'un levier de négociation qui peut être utile. Néanmoins, si les emplois concernés sont organisés en statut d'emploi, rien n'empêche le pouvoir réglementaire de prévoir l'application d'une grille de rémunération aux fonctionnaires et aux non-fonctionnaires, comme c'est aujourd'hui le cas, par exemple, pour les préfets. L'avis est donc défavorable.

Il vise à introduire deux garanties pour les contrats de droit public qui sont actuellement exigées pour les contrats de droit privé : d'une part, il fixe une durée minimum légale de travail à vingt-quatre heures pour les temps partiels ; d'autre part, il limite à deux le nombre de renouvellements de contrats à durée déterminée. Ces deux mesures participeront de la lutte contre la précarité dans la fonction publique, puisque leur efficacité est aujourd'hui reconnue dans le secteur privé.

nous considérons qu'il est possible de contourner cet obstacle des regroupements. Nous pensons surtout que le rapprochement entre le secteur privé et le secteur public doit se faire en s'alignant sur le régime le plus protecteur pour les salariés, et non pas l'inverse. Quel est l'avis de la commission commission ? Cet amendement a pour objet d'imposer une durée minimale de travail hebdomadaire pour les agents contractuels à temps partiel, dans les trois versants de la fonction publique. Elle serait fixée à vingt-quatre heures par semaine, comme c'est le cas, en principe, pour les salariés de droit privé. Je rappelle cependant qu'il existe de nombreuses dérogations à cette règle dans le secteur privé.

? Pourquoi se priver de la possibilité d'avoir un contractuel plus longtemps ? L'avis est donc défavorable.

Laurence Cohen, sur l'article. Selon les chiffres du Gouvernement, l'élargissement du recours au contrat concernerait 3 800 emplois de la fonction publique de l'État, 1 522 à 2 700 emplois de la fonction publique territoriale et 365 emplois de la fonction publique hospitalière. Cela représente une augmentation du nombre de contractuels de 456 dans la fonction publique de l'État, de 77 % dans la territoriale et de 28 % pour l'hospitalière. Alors que, depuis trois mois, les services d'urgences sont engagés dans un mouvement de grève pour alerter la population et le Gouvernement sur les conditions intolérables d'accueil et de prise en charge des patients, alors que plus de cent services d'urgences sont mobilisés, sous diverses formes, pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail, le manque de moyens, mais surtout la dégradation des soins offerts aux patients, vous allez encore, monsieur le secrétaire Alors que les personnels sont au bord de l'épuisement généralisé et que les services sont saturés- ils risquent de l'être encore plus si l'été est, comme cela est annoncé, caniculaire -, vous affaiblissez le service public et mettez en danger les patients et les personnels. Quand on rencontre les personnels hospitaliers- soignants, administratifs, ouvriers, direction -, ils nous font part de leur besoin de travailler au sein d'équipes stables, qui se connaissent et qui ont l'habitude de fonctionner ensemble. Croyez-vous vraiment que la généralisation des contrats résoudra les difficultés ? des syndicats demandent au contraire la titularisation de tous les contractuels. Que cet article se concentre sur les emplois supérieurs hospitaliers ne change rien à l'affaire. Comment peut-on assurer la continuité du service public avec l'élargissement du recours aux contrats pour les emplois de direction dans les trois versants de la fonction publique ?

que cela sert leur carrière. Nous avons là un changement de philosophie complet ! Beaucoup disent que ce projet de loi ne remet pas en question la fonction publique. Peut-être ! Mais il permet aux fameux managers d'affaiblir la fonction publique à petit feu ! En tout cas, c'est le sentiment que nous en avons. Avant, en simplifiant, on pouvait imaginer que des contractuels souhaitent devenir titulaires pour occuper des postes de direction. Maintenant, ils n'auront aucun intérêt à penser à la titularisation. Vous mettez donc à mal l'attractivité de la fonction, laquelle est déjà bien abîmée- pas de votre seul fait, je vous l'accorde. Pour évoquer ce défi d'attractivité, je vous renvoie à un forum sur l'emploi organisé par la SNCF à Paris il y a peu. Les observateurs ont indiqué que l'affluence avait été décevante, notamment en raison de la perte d'attractivité du statut de cheminot. Pour les emplois les plus qualifiés, la SNCF ne peut rivaliser en termes de salaire. Je fais mention de ces éléments pour vous montrer que les conséquences de ce projet de loi, comme nous l'avons relevé dans la discussion générale et au fil du débat, sont bien plus lourdes à terme que ce que l'on peut imaginer.

sont visés : la très grande majorité des emplois de direction au sein des trois versants, tous les emplois des établissements publics de l'État à l'exception de ceux pourvus par les personnels de recherche, les emplois de catégories B et C de la fonction publique de l'État, les emplois ne nécessitant pas une formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un corps de fonctionnaires, tous les emplois de catégorie B de la fonction publique territoriale, tous les emplois des communes de moins de 1 000 habitants et des EPCI composés de communes dont la population moyenne est inférieure à un certain seuil et tous les emplois à temps non complet

Très concrètement, il s'agit de permettre le recours à des managers du privé pour pourvoir des postes de direction, afin d'améliorer l'efficacité du service public. Je dois vous le dire, ce présupposé que le privé est toujours meilleur que le public est une insulte pour l'ensemble des fonctionnaires de notre pays et une erreur monumentale. Cet article est extrêmement grave. Il va favoriser les allers-retours de hauts fonctionnaires entre le public et le privé, le pantouflage et le rétropantouflage, qui vont avoir pour effet d'établir, comme le souligne Anicet Le Pors, ancien ministre de la fonction publique et père du statut actuel, « une confusion des finalités du public et du privé, un accroissement du risque de conflits d'intérêts et une captation de l'action publique par la finance internationale ». C'est bien de cela qu'il s'agit. D'ailleurs, je rappelle l'avis extrêmement réservé du Conseil d'État, qui « regrette en particulier que cette étude ne fournisse aucune donnée chiffrée quant au nombre de fonctionnaires en attente d'affectation ni ne présente d'éléments relatifs à l'impact possible d'un accroissement sensible du nombre d'agents contractuels occupant, dans le cadre de contrats à durée indéterminée, tous types d'emplois dans la fonction publique sur le déroulement de carrière des titulaires et sur la coexistence de ces deux catégories d'agents

Un vrai boulevard pour le secteur privé ! Un tel dispositif permettra notamment à des dirigeants d'entreprises privées d'occuper des postes de direction d'administration, de s'y constituer des réseaux d'influence avant de retourner à leurs affaires. Un système sordide, dont nos concitoyens ne veulent plus et qui nourrit la défiance envers l'administration et les pouvoirs publics. Nous voulons une administration- une haute administration surtout -exemplaire, au-dessus de tout soupçon. Cet article ouvre la boîte de Pandore, et c'est pourquoi nous en demandons la suppression.

pour les emplois de direction. Le Gouvernement invoque son souhait de construire des parcours professionnels ascensionnels pour les agents contractuels de droit public, sans jamais apporter de réponses s'agissant des conséquences attendues sur les parcours des agents titulaires du concours, qui- on l'imagine -risquent d'être, pour le coup, moins ascensionnels le Conseil d'État regrette d'ailleurs que l'étude d'impact « ne fournisse aucune donnée chiffrée quant au nombre de fonctionnaires en attente d'affectation ni ne présente d'éléments relatifs à l'impact possible d'un accroissement sensible du nombre d'agents contractuels occupant, dans le cadre de contrats à durée indéterminée, tous types d'emplois dans la fonction publique sur le déroulement de carrière des titulaires et sur la coexistence de ces deux catégories d'agents, qui seront désormais en concurrence pour l'accès aux emplois de direction ». Cette même étude d'impact donne des indications sur le nombre de postes désormais ouverts aux recrutements sur contrat passeraient de 683 à 3 800 dans la fonction publique de l'État, de 1 522 à 2 700 dans la fonction publique territoriale et de 284 à 365 dans la fonction publique hospitalière. Autant de postes sur lesquels les fonctionnaires de catégorie A se trouveront demain en concurrence avec des contractuels. La notion de carrière dans la fonction publique perd ainsi de son sens. L'agent qui, après un parcours louable, aurait été en mesure de prendre un emploi de direction sera mis en concurrence avec des personnes n'ayant aucunement la légitimité qu'il tire du concours

l'avis du Gouvernement ? Le Gouvernement ne partage pas l'ensemble des dispositions adoptées par la commission des lois sur les questions d'encadrement- j'aurai l'occasion d'y revenir -, mais nous considérons que l'article 7 est utile. D'abord, et Mme la rapporteur a terminé son propos par ce point, il permettra de diversifier les profils occupant des emplois de direction.

Mme Gréaume évoquait les risques en matière de déontologie. C'est la raison pour laquelle, après l'article 16, nous avons prévu un contrôle systématique de la déontologie à l'entrée dans la fonction publique pour les contractuels qui seraient conduits à occuper des emplois de direction. Ainsi le garde-fou est posé. Par conséquent, l'avis est défavorable sur les amendements de suppression.

Nous avons eu un débat, y compris à l'occasion de rencontres avec les rapporteurs, sur la possibilité de recruter en contrat, de manière indifférenciée, pour l'ensemble des postes des établissements publics de l'État.

que le Gouvernement présente comme un amendement de cohérence, vise à supprimer, à l'article 7, la référence aux emplois de direction des établissements publics de l'État, au motif que l'article 9 autorise déjà les établissements publics administratifs à pourvoir l'ensemble de leurs emplois par voie de contrat.

En écho à ce que vient d'indiquer Mme le rapporteur, puisque nous restreignons le champ du contrat sur les emplois de direction à l'article 9 et que le Gouvernement souhaite le faire maintenant à l'article 7,

qui veut qu'à poste égal le salaire soit égal, peu importe le statut de l'agent- fonctionnaire ou contractuel. L'amendement

Mme Maryse Carrère. Un amendement adopté en commission des lois a introduit une obligation de formation préalable pour les agents contractuels recrutés aux fonctions de directeur d'administration centrale. L'aptitude du candidat à s'adapter à l'organisation et au fonctionnement des services publics devrait, en réalité, être l'un des premiers critères de de recrutement. Il ne paraît effectivement pas concevable de recruter à de tels postes des personnes n'ayant aucune idée des sujétions particulières s'imposant au service public. Ces formations pourraient aussi se révéler contre-productives, dès lors que l'absence de moyens mis à disposition pour les organiser pourrait justifier que l'on ne recrute pas d'agents contractuels sur ces postes. Il est d'ailleurs étonnant qu'une telle disposition soit passée entre les mailles du filet de l'irrecevabilité financière.

Cette disposition risquerait d'entraîner une politisation de ces postes de direction, qui nous paraît incompatible avec les valeurs de la fonction publique. Se poserait alors la question des conditions de recrutement de ces agents, de leur rémunération et, d'une certaine façon, de la continuité du service public. Si la fonction de DGS suppose un lien de confiance entre l'exécutif local et le premier « territorial » de l'administration, ce dernier traduisant au travers de son action les desseins politiques des élus, cette fonction ne peut être confondue avec celle d'un collaborateur de cabinet,

peut notamment être pris en charge par le CNFPT et le centre de gestion dans l'attente d'une nouvelle nomination. Aussi, l'amendement vise à supprimer cette disposition.

en deux cadres d'emplois- ingénieur et ingénieur en chef -par le décret du 26 février 2016. Cette réforme du concours et de la formation des ingénieurs en chef a justement été mise en place, depuis deux ans, dans le but de recruter et de préparer des ingénieurs statutaires à des fonctions managériales et d'expertise de haut niveau.

décrédibilise les concours, et porte donc atteinte au statut de la fonction publique. Par ailleurs, les collectivités ayant recours à ce dispositif de recrutement de non-titulaires ne jouiront pas des garanties objectives offertes par le concours quant au niveau d'études, de formation et d'expertise

Mme Sylvie Vermeillet. L'article 7 abaisse les seuils au-delà desquels le recrutement contractuel sur des emplois fonctionnels est autorisé. Désormais, un seuil de 40 000 habitants serait établi de façon uniforme pour le recrutement contractuel

d'une approche professionnelle parfois différente et d'une vision complémentaire que des contractuels ont pu acquérir dans leur parcours. Un tel recrutement sur les emplois de la fonction publique territoriale est d'ailleurs souhaité par de nombreux élus.

les coups de boutoir portés au statut risquent d'être confortés par la possibilité de changer de cadres de direction au gré des alternances. Rappelons tout de même que les fonctions de direction générale doivent se distinguer de celles de collaborateurs de cabinet. L'amendement

L'abaissement de 80 000 à 40 000 habitants du seuil permettant aux collectivités de déroger au recrutement statutaire pour pourvoir les emplois fonctionnels est en contradiction avec la réforme du concours et de la formation des ingénieurs en chef, mise en place depuis deux ans

significativement le recrutement, l'évolution professionnelle et la mobilité des ingénieurs en chef issus des concours interne et externe. Par ailleurs, les collectivités ayant recours à ce dispositif de recrutement de non-titulaires ne jouiront pas des garanties objectives offertes par le concours quant au niveau d'études, de formation et d'expertise propre aux jeunes ingénieurs en chef et nécessaire à l'exercice de leurs missions.

selon une interprétation extensive du principe de libre administration des collectivités territoriales. Afin de tenter de concilier la précision requise lors de la rédaction du décret, mais également de rassurer les employeurs publics locaux sur l'effectivité de leur libre administration, nous proposons donc de rétablir la rédaction issue de l'Assemblée nationale, augmentée des mots « sous l'autorité

qui, elles, font l'objet d'une reconnaissance légale- comme les directeurs de CCAS, d'hôpital, de régie municipale ou encore de SDIS -sans que cela soulève la moindre difficulté. Par ailleurs, le bureau de l'Association des petites villes de France du mois de mars

Les termes du débat sont les suivants. D'un côté, l'édiction d'un catalogue des missions des DGS apparaît comme un facteur de sécurisation essentiel. L'incertitude en la matière est un nid à contentieux, tant en termes de légalité des décisions, au regard notamment des doutes sur l'étendue de leurs compétences, que, le cas échéant, sur le terrain de la responsabilité. De l'autre, la solution envisagée dans le projet de loi, à savoir une liste de ces missions dressée par le pouvoir réglementaire, est apparue à la commission contraire au principe de libre administration. L'amendement vise donc à concilier ces deux points de vue, aussi légitimes l'un que l'autre, en prévoyant l'élaboration d'un catalogue des missions des DGS à titre supplétif : on y aura recours uniquement en l'absence de catalogue édicté par la collectivité.

Aussi, afin de sécuriser le recours aux contractuels pour des emplois de direction, le présent amendement vise à en limiter le nombre et à en encadrer la rémunération.

J'y suis très défavorable : ce n'est pas parce que l'on abaisse de 80 000 à 40 000 habitants la population minimale des communes autorisées à pourvoir leurs emplois fonctionnels par la voie du recrutement direct qu'il faut alourdir la procédure de recrutement. Le principe d'égal accès aux emplois publics s'applique en tout état de cause, sans qu'il soit besoin de le rappeler. Le Conseil constitutionnel a jugé, s'agissant des emplois supérieurs laissés à la décision du Gouvernement, qu'il n'était pas nécessaire d'assortir ce principe de garanties procédurales particulières, sur des emplois étroitement liés à la mise en oeuvre de la politique menée par l'autorité élue et qui sont nécessairement pourvus. Il vise enfin Il vise enfin à revenir sur les clarifications apportées par la commission en ce qui concerne la nomination aux emplois de direction hospitaliers. Contrairement à ce qui est écrit dans l'objet de l'amendement, c'est la rédaction proposée par le Gouvernement qui aboutirait à transférer le pouvoir de nomination sur les emplois de direction des établissements publics de santé autres que les CHU et les CHR du président du Centre national de gestion au directeur général de l'ARS. Il serait d'ailleurs très étrange que, pour les mêmes emplois, il existe deux autorités de nomination différentes selon qu'ils sont pourvus en faisant appel à des fonctionnaires ou à des agents contractuels. L'avis est donc défavorable.

mesure. En guise de substitution, il est proposé que ces agents « s'engagent par écrit à observer les règles déontologiques s'appliquant aux agents publics au cours et à l'issue de leur contrat De deux choses l'une : soit il s'agit de règles déontologiques dont le non-respect entraînerait des sanctions disciplinaires ou pénales, auquel cas cette précision est inutile- nul n'est censé ignorer la loi - ; soit il s'agit des lignes directrices que l'on peut trouver dans les chartes de déontologie des administrations, auquel cas les conditions dans lesquelles les agents sont appelés à en prendre connaissance relèvent, au mieux, du règlement intérieur du service concerné. Je ne crois pas utile d'ajouter du droit mou au droit mou ! L'avis est défavorable.

rectifié a pour objet d'étendre à toutes les communes et à tous les EPCI à fiscalité propre la faculté de pourvoir par contrat leurs emplois de directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques. sur le principe, car elle donne toute liberté aux autorités territoriales pour nommer leurs plus proches collaborateurs. Néanmoins, je suis attachée à l'équilibre trouvé, qui rencontre l'assentiment des employeurs publics territoriaux. Nous devons aussi veiller à préserver l'attractivité des métiers de la fonction publique territoriale, en particulier des métiers d'administrateur territorial

il est proposé de rétablir l'habilitation donnée au Premier ministre pour réglementer par décret, d'une part, la procédure de recrutement sur les emplois fonctionnels des collectivités territoriales et, d'autre part, les attributions des directeurs généraux des services des collectivités territoriales et EPCI.

de département ou de région. Dans la tradition française, ces derniers sont les seuls chefs de l'administration de la collectivité. La rédaction du décret envisagé par nos collègues députés témoigne d'une grave confusion sur les rôles respectifs de l'autorité élue et de l'administration dans une collectivité territoriale comme au sein de l'État : « Sous l'autorité et le contrôle de l'autorité territoriale, le directeur général des services [ ...] dirige et coordonne l'ensemble des services, prépare et exécute [ ...] les délibérations, décisions et arrêtés de la collectivité ou de l'établissement. [ ...] Il est en outre chargé du pilotage des ressources humaines et de veiller à la bonne mise en oeuvre du dialogue social.

277 rectifié vise à fixer un quota de contractuels parmi les emplois de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux. Je n'y suis pas favorable : cette limitation n'existe pas, en l'état du droit, pour les collectivités. Le recrutement direct y est permis sur ces emplois. également à encadrer la rémunération des contractuels occupant des emplois fonctionnels, par référence aux règles relatives aux emplois de cabinet. Or ces deux types d'emplois sont de nature différente. L'article 7 prévoit déjà que les conditions d'emploi et de rémunération de ces agents seront définies par décret en Conseil d'État. Pour ces raisons, la commission

personnage important, voire essentiel, des collectivités françaises. Madame le rapporteur, je tiens à préciser que je ne suis pas sous la coupe du lobby des DGS. Bien évidemment, résoudre cet épineux problème ne signifie absolument pas remettre en cause

il est le chef des techniciens de la collectivité et participe à la mise en oeuvre du plan de mandat, en lien direct avec l'exécutif. Est-ce aux élus, demain, de réaliser les entretiens professionnels avec le directeur du CCAS, le directeur du SDIS ou le directeur des affaires culturelles, lesquels disposent d'une reconnaissance législative

Le droit pénal lui reconnaît alors un rôle de représentant : bénéficiaire d'une délégation de signature, il serait en réalité investi d'une délégation de pouvoir implicite du fait de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à l'exercice des missions qui lui sont conférées. On comprend alors la nécessité d'une clarification légale de son champ d'intervention. Enfin, comment expliquer l'invalidation d'actes de collectivités locales pour incompétence en raison de la présence du DGS en séance de commission d'appel d'offres, de commission de délégation de service public ou de Allons-nous continuer d'accepter ce type de recours ? Il nous faut voter cet amendement, lequel constitue une réponse claire à cette problématique. Je mets aux voix

Si l'article 7 élargit les possibilités de recruter des agents contractuels afin d'occuper des emplois de direction au sein de la fonction publique, le présent amendement vise à faciliter les nominations de fonctionnaires sur des emplois de direction dans la fonction publique territoriale. Il est nécessaire d'assouplir le recrutement et de permettre à des fonctionnaires talentueux de s'engager au profit des plus petites communes pour y apporter leurs compétences sans devoir être mutés dans une plus grande commune pour espérer occuper des responsabilités

n'est donc pas propre aux emplois de direction, mais à l'ensemble des catégories, dès lors qu'il y a avancement, promotion ou réussite à un concours. Le problème tient à la règle des quotas, qui fixe le nombre de personnes pouvant bénéficier d'un avancement ou d'un changement de grade.

conservateurs territoriaux de bibliothèques et aux fonctionnaires titulaires d'un emploi à un corps ou à un cadre d'emplois dont l'indice terminal est au moins égal à la hors échelle B pour pouvoir prétendre au poste de directeur général des services. Le seuil de 40 000 habitants apparaît comme plus pertinent.

fait que la notion d'intercommunalité n'a pas d'existence en droit et qu'elle pourrait aussi bien faire référence aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qu'aux syndicats de communes, cet amendement est entièrement satisfait par l'article 6 du décret du 30 décembre 1987.

Les postes spécifiques ou à profil sont une solution. Ils constituent pourtant l'exception à la règle en concernant moins de 25 000 postes, soit moins de 3 % des postes d'enseignement. La Cour des comptes souligne que leur développement, entrepris modestement depuis 2011, est « d'une ampleur insuffisante pour modifier les conditions de l'allocation des enseignants aux postes aux postes ». Il ne s'agit pas de sortir du barème, mais de comprendre qu'il n'est pas de bonne gestion des ressources humaines de ne pas sortir systématiquement de l'indifférenciation des profils des enseignants et des postes à pourvoir.

quel rapport ! Sous les fourches caudines de l'article 40, il s'agit de nous interroger collectivement sur une anomalie du droit de la fonction publique en matière de temps de travail. Ces questions sont encadrées par le droit européen, notamment pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs. Ce cadre a d'ailleurs parfois été source d'adaptation pour la gendarmerie et les sapeurs-pompiers. a également permis d'apporter des garanties fortes aux fonctionnaires, notamment au sein de l'hôpital. Une partie de ce droit n'est pas entièrement transposée en droit national. C'est le cas des règles concernant le congé annuel non pris. Le décret du 26 octobre 1984 souligne clairement que le congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. Toutefois, sous l'impulsion de la Cour de justice, le juge administratif a reconnu le droit national

disposition. Le ministre avait alors soutenu un amendement de suppression de cette mesure, nous renvoyant au débat que nous tenons aujourd'hui. Pourquoi le contrat de projet ou le contrat de mission nous paraît-il incohérent avec l'éducation nationale ? J'entends

le débat est complexe. Il me semble pour le moins gênant de le mener comme s'il s'agissait d'un sujet annexe, alors même que les concertations avec les organisations syndicales sont en cours. un tel contrat pourrait-il s'articuler ? Le retour automatique dans l'établissement d'origine de l'enseignant ayant souscrit à un contrat de mission entraînera-t-il la mutation forcée de son remplaçant ?

Quel pourrait être ce projet ? Comment évaluer son achèvement et, encore plus, sa réussite ? Allons-nous avoir droit à des contrats sur trois ans, avec l'objectif d'atteindre tel ou tel taux de réussite aux examens, au mépris des conditions d'études de l'établissement ? Tout d'abord, cette mesure viendrait aggraver les inégalités : on sait tous que, selon les établissements, il est plus facile ou difficile de faire réussir les élèves. Ensuite, elle constituerait un détournement complet de l'objectif du service public, dès lors considéré comme une entreprise de service quelconque. La parole est à Mme Laurence Cohen, Laurence Cohen, sur l'article. Cet article institue les fameux contrats de projet, pendants pour la fonction publique des contrats de chantier du secteur privé. Ces contrats, dont le champ a été élargi par la commission des lois, puisqu'ils concernent dorénavant l'ensemble des catégories A, B et C, entérinent une précarité accrue pour les contractuels qui seront ainsi engagés. Monsieur le secrétaire d'État, dans le secteur privé, ce dispositif est réservé au recrutement des ingénieurs et des Pouvez-vous nous dire en quoi un agent recruté comme brancardier ou agent de l'état civil s'inscrit dans un tel projet ? La commission a également précisé la fin de ce contrat comme étant la fin du projet, ce qui permet utilement de s'exonérer de toute référence à une fin de contrat anticipée. Une telle définition accroît la précarité subie par les agents, car ils ne pourront pas bénéficier de l'indemnité de fin de rupture à laquelle ils auraient normalement pu prétendre. pu prétendre. Pour l'heure, ce que recouvrent les notions de projet ou d'opération n'est pas non plus précisé, comme le souligne dans une interview intéressante une avocate spécialiste de la fonction publique. Elle s'interroge ainsi sur le fait que la création d'un service puisse être qualifiée de « projet En tout état de cause, elle souligne à raison les risques de conflictualité accrus devant le juge, face à une telle faiblesse de définition de ces nouveaux contrats. Il est en effet fort à craindre que l'intégralité des effectifs affectés à la réalisation du projet en question seront recrutés sous ce type de contrat, du chef de projet aux exécutants, puisque l'ensemble des catégories sont dorénavant concernées. Il s'agit d'une manière évidente de contourner la législation actuelle sur le recours aux contractuels, qui reste encadré, et les fonctionnaires. Il s'agit tout aussi clairement d'un changement de paradigme, substituant au temps long de l'action publique et à sa permanence la mission spécifique inscrite dans une durée limitée. On se situe donc dans une conception des services publics d'usage plutôt que de l'offre. Précisément pour la fonction publique territoriale, le fait que ces nouveaux contrats de projet

pour justifier l'appui de la majorité sénatoriale à cette mesure, vous affirmez que près de 80 % des élus consultés sont pour un tel dispositif. Nous trouvons l'argument un peu court, au regard des risques juridiques induits par le champ trop large de ce dispositif et par la nocivité d'un recours généralisé à ces pratiques.

besoin se fasse entendre, notamment auprès de certaines petites collectivités. Mais de là à prévoir des contrats aussi longs, hybrides et peu protecteurs, il y a un monde ... Comment justifier des différences de durée avec le privé ? Ces

symbolique de la démarche du Gouvernement, visant à rapprocher le droit de la fonction publique du droit du travail

tous les postes pourront être pourvus par ces contrats de projet, alors que, dans le privé, ils ne concernent que les postes d'ingénieur et de cadre.

il est parfois nécessaire de recruter, pour une période courte, un cadre ou une personne ayant des compétences particulières, pour accompagner

contrat de projet. Ils ne pourront eux-mêmes faire aucun projet, car, avec une telle incertitude quant à leur devenir professionnel, ils seront dans l'incapacité d'accéder à un bail ou à un prêt. Cet article est dangereux, car il réussit le tour de force de mettre en place, dans la fonction publique, un contrat d'une extrême précarité, avec lequel le travailleur ne bénéficiera ni des avantages d'un contrat de droit public ni de ceux

Il revient sur l'idée, pourtant essentielle, que le fonctionnaire est au service de l'intérêt général, responsable devant la Nation, ce qui suppose son indépendance face aux pressions économiques et politiques. C'est pour cela qu'il bénéficie d'un emploi permanent, régi par un statut et non par un contrat. Or, sous couvert de souplesse, ce qu'on nous propose au travers du développement des contrats de projet, c'est toujours plus de précarité pour les agents publics et une fragilisation des missions de service public qu'ils remplissent. Notre pays a au contraire besoin de services publics renforcés. C'est d'ailleurs le constat du dernier rapport du Défenseur des droits.

de faire grève, de s'opposer, lorsqu'un contrat risque de ne pas être renouvelé. Ce recul va de pair avec l'affaiblissement des organisations syndicales, que prépare cette réforme.

Or nous avons justement besoin de services publics renforcés, ce qui suppose des fonctionnaires expérimentés, pour répondre aux défis croissants et si complexes auxquels notre pays est confronté. Voilà pourquoi il faut assurer une gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences à long terme,

n° 118 rectifié. Édouard Philippe avait dit son soutien aux contrats de chantier, en indiquant que c'était pour lui un instrument intéressant parce qu'il maintenait le CDI comme norme. Dans la même logique, vous allez sans doute

peuvent nécessiter, pour la réalisation de missions ou de projets très spécifiques, des outils particuliers. Il faut en tenir compte. Mais le recours à des outils favorisant la précarité n'est pas, pour nous, une solution acceptable. Le contrat de projet, tel qu'il est proposé par le Gouvernement, concentre tous les facteurs de précarité. À la différence du contrat de chantier prévu à l'article L. 1223-8 du code du travail, qui est un CDI, le contrat de projet de la fonction publique est à durée déterminée. Cette qualification aurait dû donner lieu à une prime de précarité à l'issue du contrat, mais le Gouvernement a explicitement exclu les contrats de projet du bénéfice des primes de fin de contrat-

de projet est possible pour mener à bien un projet ou une opération spécifique. L'article ne conditionne pas son recours à des besoins temporaires. Pourtant, c'est au nom de ce même caractère temporaire qu'un contrat de projet ne pourra conduire ni à une CDIsation ni à une titularisation. Le contrat de projet pourra être rompu unilatéralement, si le projet se termine de manière anticipée ou ne peut pas se réaliser. Cette disposition pourra provoquer d'importants contentieux : qu'adviendra-t-il si le salarié considère que l'employeur a estimé à tort que le projet était terminé ou qu'il ne pouvait se réaliser ?

pour mener à bien un projet ou une opération identifié, recruter un agent par un contrat à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation du projet ou de l'opération ». Ce dispositif ne remet pas en cause

signataires. Ce contrat, que nous voulons à la fois souple et protecteur, s'adresse aussi à des hommes et des femmes qui, dans notre pays,

à des hommes et des femmes qui ont des compétences particulières de servir l'action publique pendant quelques années, à l'échelle d'un contrat de un à cinq ans, pour répondre aux besoins des administrations. Telle est la philosophie de ce contrat. Nous assumons

parole est à M. Didier Marie. En vertu de la rédaction actuelle de l'article 8, le recours au nouveau contrat est possible « pour mener à bien un projet ou une opération identifié ». Cette formulation, aussi large que floue, permettra de faire entrer dans le champ de ce nouveau contrat l'essentiel des contrats à durée déterminée actuels. De ce fait, les CDD aujourd'hui conclus pourraient demain être remplacés par ces contrats dits « de projet », qui, à leur terme, échappent au versement d'une prime de précarité et à la possibilité de transformation en CDI.

vise à répondre à la conduite de projets nécessitant des compétences spécifiques. À cet égard, l'étude d'impact donne plusieurs exemples d'application de contrats dits « de projet », comme la réorganisation des outils en matière de ressources humaines ou la maîtrise d'ouvrage dans un chantier complexe, qui correspondent

à M. Didier Marie. Cet amendement tend à aligner la durée minimale du contrat de projet du secteur public sur celle prévue en droit du travail pour le secteur privé, soit dix-huit

Cet amendement vise à aligner la durée maximale du contrat de projet du secteur public sur celle prévue en droit du travail pour le secteur privé, soit

Or un projet d'une durée équivalente à un mandat n'entre pas dans le champ des besoins temporaires. Nous avons eu un débat qui a suscité un peu d'émotion sur les procès qui pourraient être intentés à des employeurs recourant de manière excessive à des emplois contractuels. Le risque

afin d'assurer l'équilibre entre le besoin de flexibilité de ces employeurs et la nécessité d'accorder une sécurité minimale aux personnes recrutées par cette voie, nous proposons de mieux encadrer les conditions de résiliation prématurée de ce contrat, telles qu'elles ont été clarifiées par la commission des lois. Dans cette optique, le présent amendement tend à créer un droit de reclassement pour les agents recrutés par voie de contrat de projet lorsque ce dernier est mené à bien mené à bien avant la fin de la durée initialement prévue. Il s'agit également d'une garantie pour les employeurs, dès lors que la perspective de bénéficier d'un avenant pour travailler sur un nouveau projet permettra de s'assurer que l'agent concerné réalisera ce projet de la manière la plus efficace possible.

aux causes possibles de résiliation anticipée d'un contrat de projet, en spécifiant que celle-ci ne pourra intervenir, outre la réalisation de ce projet, que lorsqu'un évènement étranger à la volonté des parties le justifiera. La rédaction proposée ici pour encadrer les circonstances de résiliation s'inspire de la théorie jurisprudentielle de l'imprévision développée par le juge administratif. Il s'agit de s'assurer que l'employeur agira en responsabilité au moment du recrutement et de la résiliation d'un tel contrat, afin d'éviter des dépenses publiques inutiles provoquées par le fait du prince. L'article 8 du projet de loi instaure des contrats de projet pour une durée maximale de six années. Ces contrats doivent avoir pour but de mener à bien un projet ou une opération spécifique

que pour l'exercice d'une fonction requérant des qualifications spécialisées et ne pas entraîner la précarisation des agents les moins qualifiés.

en cas de vacance temporaire d'emploi dans la fonction publique territoriale qu'a décidé votre commission. Nous considérons que la fixation à deux ans, au maximum, des contrats de vacance temporaire institués par la loi Sauvadet de 2012 ménage un équilibre entre la nécessité de souplesse dont doit disposer l'employeur et la prévention de la précarité des agents contractuels. De plus, l'ouverture de la possibilité de recruter par voie de contrat sur des emplois à tous les niveaux, prévue dans le présent projet de loi, offre des souplesses qui nous paraissent

129 rectifié vise à préciser que le projet ou l'opération pour lequel serait conclu un contrat de projet doit « répondre à un besoin temporaire » et « nécessiter des compétences spécifiques

on parle d'emplois du niveau de la catégorie A, B ou C pour désigner les emplois permanents qu'ont vocation à occuper les fonctionnaires appartenant aux corps ou aux cadres d'emplois de catégorie A, B ou C. C. Surtout, par définition, les emplois créés pour mener à bien un projet ponctuel ne correspondent à aucun des emplois permanents qu'ont vocation à occuper des fonctionnaires.

A. L'amendement n° 120 rectifié vise à porter de un an à dix-huit mois la durée minimale du contrat de projet, comme c'est le cas dans le secteur privé. Le contrat ne pourrait donc être rompu par anticipation, au motif que le projet ne peut pas se réaliser,

du travail. Or cette modification serait, à mon sens, défavorable à l'agent. En effet, contrairement à un salarié de droit privé, un agent public en CDD peut toujours démissionner sans avoir à payer de dommages et intérêts à son employeur. Les conditions de licenciement sont également plus souples qu'en droit du travail, mais le licenciement doit tout de même être motivé par l'intérêt du service. C'est pourquoi j'invite nos collègues à retirer leur amendement ; à défaut, l'avis sera défavorable.

pas se réaliser, dès lors qu'une « offre » d'emploi serait publiée dans un délai de deux mois pour un projet ou une opération « comparable ». J'en comprends l'intention, mais cette rédaction donnerait

l'article 8 prévoit que, à l'expiration de la durée minimale d'un an, le contrat de projet puisse être rompu de manière anticipée par l'employeur, dans le cas où le projet ou l'opération ne peut pas se réaliser. Ce dispositif s'inspire du droit du travail, dans lequel le contrat à objet défini peut, à l'expiration de sa durée minimale de dix-huit mois, puis à la date anniversaire de sa conclusion, être rompu pour tout motif « réel et sérieux ». Il ne faut pas forcer l'analogie,

Cet amendement tend à préciser que la rupture anticipée du contrat n'est justifiée que si le projet ou l'opération ne peut pas se réaliser « du fait d'un évènement étranger à la volonté des parties ». J'y suis favorable, car cela correspond à l'intention de la commission. En dehors de ce cas, le contrat pourra toujours être rompu par anticipation, soit par la démission de l'agent, soit par son licenciement, dans les conditions du droit commun. Concernant l'amendement n°

ils sont satisfaits, car la réglementation applicable aux positions des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales autorise déjà leur détachement sur contrat. Je vous renvoie, pour la fonction publique de l'État, à l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 et, pour la fonction publique territoriale, à l'article 2 du décret du 13 janvier 1986. Les conditions du détachement mériteraient sans doute d'être assouplies dans la fonction publique hospitalière, mais cela relève

Les employeurs publics locaux peuvent avoir recours à un agent contractuel pour faire face à une vacance d'emploi, dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée maximale d'un an, sa durée peut être prolongée jusqu'à deux ans, lorsque la procédure de recrutement d'un fonctionnaire n'a pu aboutir. Sur l'initiative de plusieurs de nos collègues, la commission a porté cette durée maximale à trois ans,

par de nouvelles souplesses, vouloir leur opposer l'exigence que le statut soit la seule modalité

à recourir à des marchés avec des prestataires, pour réaliser en interne des projets, par le moyen du contrat de projet. Je ne vois pas en quoi ce pourrait créer de la précarité, alors qu'il crée, au contraire, de l'emploi public qui n'existait pas, et je ne vois pas en quoi il porterait atteinte aux Tables de la Loi d'un statut qui a été conçu, je le répète,

l'amendement n° 25. Dans le prolongement des articles précédents, l'article 9 étend le recours aux contractuels sur des postes permanents de la fonction publique de l'État ainsi que dans des établissements publics administratifs, en lieu et place du recrutement par concours et de l'application du statut. Or, vous le savez parfaitement, le concours et le statut permettent de garantir l'impartialité et l'égalité de traitement. Le concours répond à des exigences, pourtant évidentes, tenant à la notion même d'État, qui ne doit exprimer ni faveur ni préférence, qui ne peut discriminer et qui ne doit tenir compte que des compétences et du mérite des candidates et candidats. Les fonctionnaires titulaires ne sont pas des salariés, mais des serviteurs de l'État.

secrétaire d'État, vous ouvrez les vannes d'un recrutement clientéliste, politique ou relationnel. Bref, vous privatisez la fonction publique de l'État. Si nous partageons les conclusions du rapporteur, qui souligne que « l'extension du recours au contrat à tous les emplois des établissements publics administratifs administratifs de l'État [ ...] est dangereuse » et pourrait renforcer le démembrement de l'État auquel « il doit être mis fin », nous pensons, toutefois, que c'est sur toute extension de la contractualisation qu'il aurait fallu revenir. En effet, l'application au secteur public de méthodes de gestion traditionnellement réservées au secteur privé est incompatible avec la préservation de l'intérêt général et la satisfaction des usagers. On ne peut répondre aux attentes de nos concitoyens à moindre coût, mais c'est pourtant là toute la philosophie du nouveau management public que vous déclinez dans ce projet de loi, sous couvert du triptyque économie, efficacité, efficience. Le nouveau monde ressemble étrangement à un vieux dogme

Pour rappel, le recours aux agents contractuels est une dérogation au principe selon lequel les emplois permanents doivent être occupés par des fonctionnaires. Actuellement, il est possible, pour un employeur public d'État, de recruter des contractuels sur des postes permanents pour les seuls emplois de catégorie A et si la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Par cet article, cette faculté serait étendue aux emplois de catégories B et C, selon des critères élargis. Ce recrutement par contrat serait toujours possible lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, comme le prévoit le droit en vigueur, mais l'article précise ces conditions pour leur donner une portée plus large que celle que leur confère la jurisprudence administrative.

Concernant les besoins du service, l'article assouplit le critère pour l'employeur, puisque le candidat fonctionnaire devra présenter l'expertise ou l'expérience professionnelle adaptée aux missions à accomplir. Il suffira donc pour l'employeur de considérer que tel n'est pas le cas pour pouvoir recourir au recrutement par contrat. Enfin, l'article ajoute une hypothèse supplémentaire de recours aux contrats lorsque l'emploi ne nécessite pas une formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un corps de fonctionnaires. Ces dispositions sont élargies aux établissements publics de l'État. L'objectif est toujours le même : mettre en concurrence les fonctionnaires avec des contractuels et réduire la portée du statut,

la commission ? L'article 9 étend les possibilités de recours aux agents contractuels dans la fonction publique de l'État. La commission l'a ramené à des proportions plus raisonnables : il s'agit seulement que des emplois permanents de toute catégorie puissent être occupés par des contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, c'est-à-dire lorsque l'administration n'est pas en mesure de faire appel à un fonctionnaire. Dans ces conditions, nous sommes défavorables à sa suppression. Quel est

les lignes de conduite qui sont les nôtres. Par ailleurs, j'aurai l'occasion dans un instant de présenter des amendements de rétablissement de certaines dispositions que la commission des lois du Sénat a supprimées, afin de restreindre l'ouverture de cette possibilité de recours aux contrats ; le Gouvernement souhaite,

il s'agit d'étendre la dérogation dont bénéficient aujourd'hui plus d'une vingtaine d'établissements publics à l'ensemble des établissements publics de l'État, qui pourront ainsi recruter, en fonction de leurs besoins, la compétence souhaitée.

l'existence d'un principe à valeur constitutionnelle qui interdirait de différencier les règles applicables au recrutement d'agents publics dans les établissements publics. En tout état de cause, la procédure que nous prévoyons à l'article 6 s'appliquerait à ces établissements. amendement tend à rétablir l'une des conditions du recrutement infructueux en cas de vacances d'emploi. Les besoins du service impliquent que l'autorité de recrutement ne soit pas en mesure de pourvoir l'emploi ne soit pas en mesure de pourvoir l'emploi par un fonctionnaire présentant l'expertise ou l'expérience professionnelle adaptée aux missions à accomplir à l'issue du délai prévu par la procédure mentionnée à l'article 61. L'amendement n° 384, présenté par le Gouvernement, Cet amendement vise à rétablir la possibilité de recruter par voie de contrat, lorsque l'emploi ne nécessite pas une formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un corps de fonctionnaires. Il s'agit d'une souplesse nouvelle accordée aux employeurs de l'État, dans le respect du principe d'occupation des emplois permanents par des fonctionnaires. Elle nous permettra d'élargir de manière importante les viviers de recrutement et de mieux répondre aux besoins exprimés par les services. Quel est l'avis de la commission

? L'amendement n° 374 vise à rétablir une disposition supprimée en commission, qui permettrait aux établissements publics administratifs de l'État de pourvoir l'ensemble de leurs emplois par voie de contrat. Aujourd'hui, une vingtaine d'établissements publics, énumérés par décret, ont la faculté de recruter des agents contractuels sur des emplois qui requièrent des qualifications particulières indispensables à l'exercice de leur mission spécifique et non dévolues à des corps de fonctionnaires, en application du 2° de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984. Par exemple, l'Agence française pour la biodiversité peut recruter des agents contractuels sur des emplois de catégorie A requérant des qualifications particulières en matière d'écotoxicologie, de chimie des milieux aquatiques ou de pollution diffuse. diffuse. Le musée du Quai Branly dispose de la même faculté pour des emplois de catégorie A nécessitant des qualifications particulières, comme ceux de commissaire d'exposition, d'organisateur d'évènements, de régisseur, de restaurateur et de responsable de collection en art extra-occidental. Ces dispositions dérogatoires, qui s'expliquent par la forte spécificité des missions exercées par les établissements publics concernés, se justifient parfaitement. En revanche, l'amendement est adopté, n'importe quel emploi de n'importe quel établissement public administratif pourra être pourvu par voie de contrat, même lorsqu'il existe des corps de fonctionnaires d'État parfaitement à même de remplir ces fonctions. Cette évolution nous paraît dangereuse : elle conduirait inévitablement à la multiplication des créations d'établissement public, c'est-à-dire à la poursuite du démembrement de l'État, à la seule fin de contourner les règles de recrutement auxquelles l'État est astreint. Elle est en outre illégitime, car, même si certains établissements publics exercent des missions très spécifiques, ce n'est pas nécessairement le cas. Un établissement public administratif n'est qu'un service public administratif auquel il a été décidé de donner la personnalité juridique. le Conseil d'État a rappelé qu'un principe de parité devait continuer à s'appliquer en la matière entre les services personnalisés et les autres. Enfin, Enfin, l'argument tiré de l'autonomie des établissements publics est assez curieux : un établissement public est certes soustrait à la hiérarchie administrative de droit commun, mais pas à toute tutelle ; surtout, il n'est pas au-dessus des lois, non plus d'ailleurs que les collectivités territoriales, dont l'autonomie est constitutionnellement protégée. L'avis est donc défavorable

il vise à rétablir une disposition supprimée en commission, en vertu de laquelle les administrations de l'État pourraient pourvoir par voie de contrat tous les emplois ne nécessitant pas de formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un corps de fonctionnaires.

Nous proposons de permettre la création dans la fonction publique hospitalière d'un contrat pour besoins saisonniers, sur le modèle du dispositif en vigueur dans la fonction publique de l'État et la fonction publique territoriale, de manière à pouvoir satisfaire des besoins ponctuels et saisonniers. Il s'agit d'une harmonisation entre les trois versants

Alors que la crise est patente dans la fonction publique hospitalière, le Gouvernement invente des saisonniers

et voter comme un seul homme

que nul n'est capable de dire si la personne qui le reçoit au guichet d'un hôtel de ville, de la sécurité sociale ou d'un hôpital est titulaire ou contractuelle. Chaque fois qu'on utilise des mots comme « nocivité », « mercenaires », d'autres que j'ai entendus dans d'autres

est à M. le secrétaire d'État. Cet amendement vise à permettre aux établissements d'enseignement supérieur de recruter des salariés de droit privé dans leurs exploitations agricoles et dans les centres hospitaliers universitaires vétérinaires et à soumettre ces agents aux dispositions du code du travail et du code rural et de la pêche maritime. Cette disposition existe pour les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole, en application du code rural et de la pêche maritime.

et du travail administratif sont peu compatibles avec des missions très particulières, notamment de soins prodigués ou de traite des vaches le matin et le soir, week-ends compris ; je pense aussi aux amplitudes horaires importantes

les centres hospitaliers universitaires vétérinaires que comprennent ces établissements d'enseignement supérieur. Il s'agirait des ouvriers agricoles travaillant dans les exploitations pédagogiques et des praticiens hospitaliers officiant dans les CHUV. Nous pouvons entendre l'argument du Gouvernement selon lequel, pour ses agents issus du secteur privé, où ils sont couverts par des conventions collectives, il est préférable d'éviter toute rupture de régime social et de retraite, en les maintenant sous un régime de droit privé.

Encourager la diversité des viviers de recrutement, objectif invoqué dans l'exposé des motifs, ne passe pas, à nos yeux, par un contournement du concours, mais par une refonte des concours pour qu'ils répondent mieux au besoin de diversité au sein de la fonction publique. Nous considérons que les fonctionnaires restent, hormis pour des missions très spécifiques, les mieux à même, de par la construction républicaine de leur statut, de faire face à des missions particulières, qui relèvent de l'intérêt général. C'est d'ailleurs la nature de ces missions si spécifiques qui a conduit les fondateurs du statut à soumettre les fonctionnaires à un ensemble de devoirs et de droits qui leur permettent d'assurer l'égal accès de tous aux services publics.

à l'ensemble des catégories, lorsque les besoins du service ou la nature des missions le justifient. Cet élargissement est bien trop large et permettra un recours massif aux contractuels.

soit plus de 4 500 communes de plus que ce que prévoyait le projet de loi initial, pourront recourir au contrat pour l'ensemble de leurs agents. Nous demandons la suppression de cet article, qui organise le dépérissement de la fonction publique territoriale, engageant un changement profond de la nature de l'action publique territoriale et sa captation par le privé. Menacer la fonction publique territoriale correspond à nos yeux à une rupture franche avec l'égal accès de tous aux services publics et avec l'égalité républicaine. Cette démarche accompagne parfaitement le projet présidentiel de suppression de 50 000 postes dans la fonction publique territoriale, en substituant aux fonctionnaires des contractuels précaires, aux droits limités et aux missions déconnectées de l'intérêt général. Quel la commission ? Nous sommes défavorables à la suppression de cet article, qui a pour objet principal d'assouplir, dans des limites raisonnables, les conditions de recrutement d'agents contractuels dans la fonction publique territoriale. Quel est l'avis du

mémoire courte : les contractuels sont entrés massivement dans la fonction publique en 1981, sur ordre, pour recruter ! On peut aussi s'interroger sur les effets de la loi Le Pors, heureusement corrigés par la loi Sauvadet pour aider